l'OMS ajoutait que « l'obésité infantile et le marketing des produits peu sains font partie des sujets de préoccupation majeurs », et que « le marketing digital pour ces produits est un nouveau défi

en sel ou en matières grasses. Seraient exemptés de cette interdiction les produits de qualité labellisés, afin- bien évidemment -de ne pas pénaliser les produits de nos terroirs. Les mentions obligatoires prévues à l'article 2 C pour intégrer une information à caractère sanitaire dans la promotion de ces produits de mauvaise qualité nutritionnelle semblaient déjà insuffisantes- elles ont d'ailleurs été supprimées en commission. Une interdiction stricte apparaît d'autant plus nécessaire. Face à l'arsenal de communication des industries agroalimentaires, les pouvoirs publics ne se battent pas à armes égales.

Des travaux scientifiques montrent ainsi que la consommation d'aliments de mauvaise qualité nutritionnelle augmente de 61 % les risques de maladies cardiovasculaires, de 40 % le syndrome métabolique et de plus de 60 % le risque d'obésité chez l'homme. Toutes ces maladies chroniques coûtent plus de 55 milliards d'euros par an, alors que le chiffre d'affaires annuel de l'agroalimentaire est de 166 milliards d'euros. On voit bien que se pose ici une question de santé publique,

La question du marketing et de la publicité ciblant les enfants sur les réseaux sociaux mérite qu'on en mesure bien les effets en matière de santé publique, d'autant que les mécanismes d'autorégulation fonctionnent mal sur ces médias. Or, à l'âge de 11 ans, plus de la moitié des enfants sont déjà présents sur les plateformes des réseaux sociaux ; ce taux passe à plus de 70 % pour les adolescents à partir de 12 ans. Les jeunes sont exposés à une grande quantité de contenus publicitaires promus par les influenceurs pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Ces boissons et aliments contribuent fortement au développement de l'obésité et favorisent des maladies chroniques comme le diabète de type 2 ou encore certains cancers. En France, un enfant sur six est en surpoids ou obèse et risque de le rester à l'âge adulte.

à interdire explicitement la promotion par les influenceurs de boissons et produits alimentaires trop sucrés, trop gras ou trop salés à destination des enfants de moins de 16 ans.

augmentation de la consommation d'alcool chez les adolescents et les jeunes adultes. Si la publicité pour l'alcool a été autorisée sur les services de communication en ligne en 2009, c'était avant l'apparition d'Instagram, de Snapchat ou encore de TikTok, plateformes utilisées le plus souvent par les mineurs. Il convient donc d'adapter la loi Évin, qui avait pour objet de renforcer la protection de la santé des jeunes. Les mineurs sont largement confrontés à ces publicités. L'association Addictions France a d'ailleurs relevé en dix-huit plusieurs milliers de contenus en faveur de l'alcool, émis par des influenceurs. Cet amendement vise à mettre en place un système en ligne permettant d'exclure l'audience mineure des publicités pour l'alcool sur le modèle de ce qui est prévu pour les jeux d'argent et de hasard à l'article 2 B de la présente

une rupture d'égalité qui n'est pas justifiée. Les amendements n 43 et 10 visent à renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de seuils à partir desquels des boissons et produits alimentaires

L'amendement n 26 rectifié vise à appliquer à la promotion de boissons alcooliques ainsi qu'à celle de boissons non alcooliques, mais commercialisées sous le nom d'une marque d'alcool, l'encadrement prévu pour la promotion des jeux d'argent et de hasard, à savoir leur autorisation sur les seules plateformes en ligne

vous le savez, la loi Évin autorise la publicité pour l'alcool sur les services de communication en ligne, dont les réseaux sociaux. La commission s'est exprimée en faveur du maintien du cadre légal existant, car l'objet de cette proposition de loi n'est pas de faire évoluer la loi Évin, loi Évin, mais de faire respecter les règles existantes et de mieux les faire connaître. Pour faciliter le travail de régulation des contenus frauduleux, la commission a attribué aux associations luttant contre l'alcoolisme, telles qu'Addictions France, le statut de signaleurs de confiance

malbouffe qui détruit la santé de nombreuses personnes qui resteront dans cet état pendant des années et des années. On peut toujours dire qu'il n'y a pas d'épidémie d'obésité, les statistiques sont très claires

Cet amendement tend à étendre l'interdiction de la promotion directe ou indirecte de produits, actes ou prestations contre rémunération aux produits paramédicaux ayant un effet amincissant supposé. Entre notamment dans le champ de cette interdiction la promotion de crèmes, de pilules ou encore de thés amincissants. La promotion de ces produits contribue en effet à propager des stéréotypes sexistes sur le corps des femmes et des hommes et peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé mentale et physique des adolescents. Cette injonction à la maigreur, très présente sur les réseaux sociaux, engendre une pression qui peut être difficile à gérer pour des jeunes en pleine construction, dans une période de grande vulnérabilité quant à l'estime de soi et surtout quant à

au culte du corps sur les réseaux sociaux. Bien entendu, tout cela est multifactoriel. Je ne dis pas que seuls les influenceurs sont responsables de ce culte de l'image ; celui-ci est présent partout dans notre société.

en rendant applicable le régime de sanctions pénales pour des infractions similaires déjà prévu par l'article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure. Quel

les effets : dépression, anxiété, culpabilité, solitude, isolement, perte d'estime de soi, parfois même le suicide. Ces jeux de hasard et d'argent ont donc un impact bien réel sur la vie des gens,

informatif pour les jeux d'argent et de hasard. Elle oblige aussi à réserver la promotion de ces pratiques aux seules plateformes permettant d'exclure effectivement les mineurs. Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Toutefois, elles se concentrent presque exclusivement sur les mineurs. Si cette population vulnérable, influençable, doit être protégée, nous souhaitons aussi protéger

Cet amendement ne perturberait pas l'écosystème économique des influenceurs, mais aurait un impact réel sur la protection de leur public face à des pratiques particulièrement nocives. La parole

avons réussi à la maintenir étanche. Mais voilà qu'un certain nombre de jeux vidéo prennent la forme de jeux d'argent- et que des jeux d'argent prennent la forme de jeux vidéo. Cela induit

dont on connaît le pouvoir de conviction sur ces consommateurs. Il nous semble donc très important d'opérer une distinction entre le jeu vidéo et le jeu d'argent qui se camoufle sous un jeu vidéo. Certes, il y a des opportunités de développement technologique, avec des réussites commerciales possibles, et de belles entreprises cherchent à se développer dans notre pays. Mais tenir les enfants et les plus jeunes à distance du jeu d'argent me paraît nécessaire à la fois pour ces personnes et pour le jeu vidéo lui-même.

aux obligations relatives aux jeux d'argent et de hasard définies à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure. Cette assimilation est contradictoire avec l'objectif de sécuriser le développement du jeu vidéo. Par ailleurs, le Gouvernement proposera au Parlement des dispositions en ce sens

et nous sommes heureux que la France puisse être considérée comme un leader dans le secteur. Mais cette ambiguïté ne bénéficiera pas aux jeux vidéo et elle n'est pas à l'honneur de ceux qui avancent masqués. Je n'ai pas envie d'interdire telle ou telle politique et je pense que l'amendement qui avait été adopté la semaine dernière en commission aurait pu être soutenu par le Gouvernement. En quoi ceux qui développent des jeux qui sont à la frontière des jeux d'argent auraient-ils besoin de faire de l'influence auprès des mineurs ? Je pense vraiment qu'il faut conserver le dispositif voté la semaine dernière, en le modifiant pour adapter la législation le moment venu. Alors que tout le monde veut protéger les mineurs sur internet, il paraît curieux que nous tergiversions ce soir ...

en plus du blocage de la promotion de produits et services interdits aux mineurs. Le présent amendement vise également à interdire la promotion de ces produits et services par des mineurs, en particulier des mineurs de 16 et 18 ans. On peut penser en particulier aux paris sportifs, qui comportent de vrais risques d'addiction et sont normalement interdits aux mineurs.

du III de l'article 2 B, un régime de sanctions adapté, en rendant applicable le régime de sanctions pénales pour des infractions similaires prévu par l'article L.

Je vous propose d'adopter l'amendement n° 81, qui fait figure de compromis puisqu'il maintient, par principe, le régime de sanctions adopté en commission, sous réserve des sanctions déjà prévues par le code de la consommation et par le code de la sécurité intérieure.

Cette disposition permettrait également d'inciter les influenceurs à adopter des pratiques respectueuses de la loi. S'il est vrai que le juge peut déjà ordonner à un opérateur condamné en raison de certains manquements de communiquer sur cette condamnation par tout moyen, tiers, par exemple le fournisseur de services de communication publique, de publier la condamnation en cas de carence, nous pensons que notre amendement aura un effet de sensibilisation plus fort. Quel

La DGCCRF a annoncé la semaine dernière qu'une première liste de trente influenceurs condamnés pour des infractions au code de la consommation serait rendue publique. Si les infractions sont bien commises à titre individuel, l'objectif de cette proposition de loi est d'encadrer une activité commerciale avant de sanctionner les individus. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable

les influenceurs s'appuient sur des contenus divers, qui mobilisent souvent des oeuvres créées par d'autres. Si les réseaux sociaux ont développé des outils pour protéger certains artistes, comme les compositeurs et musiciens-interprètes, d'autres oeuvres y sont moins bien protégées.

L'article 2 de cette proposition de loi précise que le respect du droit de la propriété intellectuelle figure parmi les obligations des parties prenantes au contrat d'influence commerciale. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable. Quel est

L'affluence et la concentration de touristes sur des sites naturels fragiles inquiètent leurs gestionnaires, qui appellent à un renforcement des moyens de régulation de ces flux touristiques. L'identification de ces sites dans des contenus postés en ligne par des utilisateurs très suivis sur les réseaux sociaux renforce les flux en question, exposant la faune et la flore qui s'y trouvent. C'est particulièrement le cas des littoraux.

Ils disposent ainsi du droit d'appliquer une redevance aux équipes de tournage qui se rendent sur ces sites et peuvent leur imposer des protocoles très contraignants d'accès aux lieux, afin de protéger les espèces qui s'y trouvent. Les conséquences de l'influence constituent un nouveau défi. C'est pourquoi je vous C'est pourquoi je vous propose de leur permettre de s'opposer aux publications d'influenceurs commerciaux mentionnant les sites dont ils ont la gestion. La surfréquentation des espaces naturels protégés est bien sûr un véritable enjeu. Le lien avec les influenceurs n'est pas évident ni avéré.

l'enfant attestait que « des données incontestables montrent que la commercialisation d'aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien direct avec l'obésité de l'enfant ». Dans un autre rapport, l'OMS ajoutait que « l'obésité infantile et le marketing des produits peu sains font partie des sujets de préoccupation majeurs

Le lien entre marketing et préférences alimentaires pour ce type de produits est aujourd'hui clairement établi. « Les enfants sont en effet particulièrement vulnérables au marketing alimentaire », lit-on aussi dans ce rapport. Afin de lutter contre l'obésité et de protéger la santé des enfants,

Notre objectif n'est pas de surréglementer l'activité des influenceurs, mais d'éviter de passer à côté d'un gros problème de santé publique. Les publicités qui visent quotidiennement les enfants sur les réseaux sociaux ne sont toujours pas responsables. L'autorégulation, d'ailleurs, ne fonctionne pas sur les réseaux sociaux. Eh oui, mes chers collègues, concurrence pure et parfaite ne fonctionne pas sur les réseaux sociaux : prenons-en acte ! Notre responsabilité est d'interdire cette publicité qui fait appel à des enfants pour mieux toucher sa cible. Il s'agit de protéger ce jeune public, plus vulnérable et particulièrement exposé à l'influence commerciale en ligne. La question n'est pas de savoir si des influenceurs peuvent, ou non, faire la promotion du lait, comme on nous l'a dit en commission pour justifier la suppression article. Mes chers collègues, le marketing pour la malbouffe matraque essentiellement les enfants, de plus en plus tôt et de plus en plus fort. D'ailleurs, dans son rapport remis au ministre de la santé le 28 avril dernier, Martine Laville rappelle que l'obésité touche surtout les enfants défavorisés. Elle est un marqueur des inégalités sociales liées à la pauvreté et au manque d'éducation. Si l'on supprime l'obésité infantile, on supprime 40 % de l'obésité tout court ! Je le répète, notre amendement vise juste- juste ! -à encadrer quelque peu la publicité pour les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés par les enfants, ciblant des enfants. Il tend à rétablir, tout simplement, l'article 2 CA voté à l'Assemblée nationale, en y ajoutant les ajustements que la rapporteure aurait proposés si l'article n'avait pas été supprimé. Les trois

fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel. Il est avéré qu'une surconsommation de boissons et d'aliments industriels, notamment de produits ultra-transformés trop sucrés, favorise la survenance

Pour lutter contre ce fléau social, l'OMS, l'OCDE et la Commission européenne ne cessent de recommander l'encadrement et la limitation du marketing alimentaire auquel sont soumis les enfants. Ce marketing évolue naturellement et trouve une nouvelle prospérité à travers les technologies du numérique et les réseaux sociaux,

d'aliments transformés ou de boissons sucrées crée un lien attractif fort avec leur jeune public, qui est ainsi incité, pour ne pas dire conditionné, à la consommation de ces produits. Pour éviter cela, l'Assemblée nationale avait- opportunément, me semble-t-il -décidé d'interdire ce type de promotion dans un nouvel article 2 CA,

que mon collègue François Bonhomme. Le marketing de ces produits est très agressif : leurs emballages sont attrayants pour les jeunes enfants, ils sont très pratiques et leurs prix sont très abordables. Nous devons absolument endiguer ce que l'OMS nomme « épidémie d'obésité et de surpoids ». La hausse de la prévalence du surpoids et de l'obésité en France est colossale. Elle est responsable de 11 % de décès supplémentaires et de 6 % des pertes d'années de vie en bonne santé, toutes

Fabien Gay, pour explication de vote. Je vais essayer d'apaiser l'hémicycle.

le temps ce qu'il ne faudrait pas faire, et que ceux qui nous donnent des leçons sont ceux-là mêmes qui proposent la dépénalisation du cannabis ! À un moment donné, il faut arrêter avec tout

15 est complémentaire à la modification introduite lors de l'examen du texte en commission concernant les obligations d'information des influenceurs en matière de formation professionnelle. de préciser les informations obligatoires à apposer par l'influenceur sur sa publication lorsqu'il effectue des communications relatives à la formation professionnelle, en complément de la mention « publicité » déjà prévue au premier alinéa de l'article 2 C. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable. Je mets

C'est la raison pour laquelle le présent amendement tend à les supprimer. Rien ne justifie d'assujettir ce type d'opération promotionnelle à des exigences particulières, dès lors que les dispositions du code de la consommation interdisent les pratiques commerciales trompeuses. Elles incluent notamment l'omission d'une information substantielle se rapportant à un bien ou à un service et imposent de fournir au consommateur, préalablement à la conclusion d'un contrat à distance,

relative à l'encadrement des promotions portant sur la souscription à un contrat d'abonnement a fait l'objet d'un consensus la proposition de loi en commission des affaires économiques. Les souscriptions à des contrats d'abonnement sont source d'escroqueries et, dans tous les cas, manquent de transparence. Ne pas savoir

Cet amendement a pour objet de rétablir le dispositif qui prévoit l'encadrement de la promotion, par les influenceurs, de denrées, de produits alimentaires et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse. À défaut d'une interdiction de la promotion de ces produits, particulièrement nocifs pour la santé de nos concitoyens- comme nous l'avons déjà dit -, le rétablissement de cet encadrement constitue un minimum. Des chiffres édifiants sur les ravages de l'obésité ont été rappelés tout à l'heure. Il faut agir, sans tarder. Le coût global de la malbouffe dépasse les 50 milliards d'euros par an, celui du diabète de type 2 représentant à lui seul 19 milliards d'euros. Pour la santé publique et l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, une politique de prévention plus ambitieuse est indispensable, comme le recommandent l'Agence Par ailleurs, ce dispositif cible uniquement les produits agro-industriels néfastes pour la santé. Leur promotion par des influenceurs doit s'accompagner, au minimum, du Nutri-score ou d'une alerte sanitaire, comme pour toute autre publicité, même si un consensus scientifique existe pour dire que ces mentions ne suffisent pas à provoquer un changement de comportement. Le choix sera donc laissé à l'influenceur entre ces deux options afin de tenir compte des caractéristiques particulières des différentes typologies de produits. La

pour la promotion de certains produits agroalimentaires. Le dispositif adopté propose de laisser aux influenceurs le choix d'ajouter à leurs publications les informations à caractère sanitaire ou le Nutri-score des produits promus. Ne sont pas concernés par cette obligation les produits labellisés,

qui demandent le renforcement des mesures de prévention. Les publicités pour les produits alimentaires sont accompagnées d'un slogan sanitaire, que nous avons pu voir, par exemple, dans les publicités télévisuelles : « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Que les influenceurs relaient ces informations de prévention dans leurs contenus promotionnels paraît être le minimum que nous puissions demander. La parole est à M.

cela a été dit à plusieurs reprises, l'article 2 A de la proposition de loi rappelle déjà le cadre juridique en vigueur en matière d'encadrement de la promotion des produits alimentaires. Vous parlez du Nutri-score. Il est à noter que les dispositions votées à l'Assemblée nationale sont moins-disantes que le droit existant, car elles laissent aux influenceurs le choix d'afficher soit le Nutri-score, soit le message d'information à caractère sanitaire, alors que ce message est obligatoire pour les promotions diffusées sur les autres canaux publicitaires. Il y a donc là

pesant sur l'influence commerciale par rapport aux canaux publicitaires par l'exemption des produits de qualité labellisés de l'obligation de délivrer un message à caractère sanitaire nous pourrions introduire une disposition contraire au droit européen, lequel impose

mais elle a généré des abus et de nombreuses arnaques. Les adaptations proposées à l'article 2 E sont donc essentielles. Toutefois, le fait de s'assurer de la disponibilité du produit pose question : des entreprises, notamment dans le textile, déclenchent la fabrication de leurs produits au-delà d'un certain seuil de commande, répondant ainsi aux préoccupations de surproduction et de consommation durable. Il est ainsi proposé de

Il est aussi tenu, toujours en tant que vendeur à distance, de respecter ce délai de livraison et il est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat, y compris lorsque la livraison est assurée par un fournisseur tiers- cela est prévu à l'article L. 221-15 du code de la consommation.

le même que celui qui est délivré aux agences de mannequinat. Nous souhaitons que les mineurs influenceurs soient accompagnés par des personnes, dont la responsabilité aura été établie par un agrément d'État

En l'état actuel du droit, les annonceurs qui souhaitent travailler avec des influenceurs de moins de 16 ans doivent signer avec eux un contrat auprès d'une agence de mannequins, et non auprès d'une agence d'influenceurs. L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence indirecte et indésirable d'autoriser les agences d'influenceurs à travailler avec des enfants de moins de 16 ans. Il existe déjà un cadre légal particulièrement protecteur pour les influenceurs de moins de 16 ans : c'est la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants L'article 1 de cette proposition de loi élargit par ailleurs le champ d'application de cette loi à toutes les plateformes en ligne, et non plus seulement aux plateformes de partage de vidéos, ce qui rendra

que la protection des mineurs est déjà assurée par les dispositions du code du travail qui encadrent l'emploi des enfants. Cet emploi est soumis à un régime d'agrément des employeurs, accordé par l'autorité administrative. proche, sans lui être identique, de celui qui s'applique aux agences de mannequins, auquel votre amendement renvoie à raison. Il convient par ailleurs de ne pas entretenir de confusion entre l'activité d'agence de mannequins et celle d'agence d'influenceurs, en particulier en raison de la différence de statut entre ces deux activités

la signature d'un contrat écrit entre l'influenceur et son agence, même lorsqu'aucune rémunération en argent n'est versée, car il peut toujours y avoir des rémunérations en nature qui ne sont pas déclarées et tous les cas doivent être envisagés. Il est donc proposé d'imposer un contrat écrit, que ce soit pour une rémunération pécuniaire ou un avantage en nature, dont le montant serait fixé par décret, afin d'éviter toute influence cachée. Quel est l'avis de la commission ? Les définitions de l'activité d'influence commerciale et d'agent d'influenceur précisent que ces deux activités s'exercent à titre onéreux. Cela inclut les rémunérations pécuniaires, mais aussi les bénéfices économiques ou les avantages en nature que les personnes peuvent retirer de ces deux activités. Par conséquent, les clauses contractuelles obligatoires précisent bien que la contrepartie perçue par les parties au contrat peut être en numéraire ou en avantage en nature. Cet amendement est donc déjà satisfait sur ce point. Par ailleurs, la commission a supprimé l'introduction d'un seuil, en somme ou en valeur, à partir duquel l'obligation de recourir à un contrat écrit s'appliquerait. C'est l'ensemble du secteur de l'influence commerciale qui doit se professionnaliser et se structurer.

est à Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de conforter les dispositions adoptées en commission et visant à faciliter l'identification des influenceurs résidant en dehors de l'Union européenne-

le statut d'entrepreneur individuel ou d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Les influenceurs installés à l'étranger doivent impérativement être rattachés à cette proposition de loi et respecter ses dispositions à partir du moment où leurs publications visent un public établi en France, ce qui est très souvent le cas, puisque leur notoriété s'est construite auprès du public français. Les personnes désignées pour assurer une représentation légale doivent ainsi être dotées de pouvoirs et de moyens suffisants afin de pouvoir coopérer, en cas de besoin, de façon efficace avec les autorités administratives et judiciaires compétentes pour assurer le respect des dispositions

l'amélioration rédactionnelle proposée par le Gouvernement, tout en s'assurant que la licéité des contenus signalés sur les plateformes s'apprécie aussi au regard des règles applicables aux influenceurs, mais pas seulement. Tous les autres contenus illicites, par exemple ceux qui diffusent des propos haineux ou de fausses informations, sont concernés par ces mécanismes de signalement. Ce n'est donc pas exclusif. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°

3 a pour objet de renforcer la responsabilisation des fournisseurs de services d'hébergement contre la diffusion de contenus illicites. Conformément au DSA, les opérateurs de plateforme en ligne devront établir des mécanismes de signalement des contenus manifestement Devant la masse des contenus à surveiller, ce mécanisme de signalement est essentiel, mais il nous semble que la responsabilité des opérateurs de plateforme en ligne pourrait aller plus loin. proposons donc de compléter le dispositif de signalement par la mise en place d'un mécanisme de suspension temporaire des comptes d'influenceurs en cas de signalements répétés de contenus illicites diffusés sur ces comptes. La suspension du compte constituerait une réponse graduée pour lutter contre les contenus illicites et contribuerait

de la responsabilité de chaque plateforme de suspendre les comptes d'influenceurs assurant la promotion de contenus illicites et faisant l'objet d'injonction de la part des autorités administratives ou judiciaires ou de signalements de la part de signaleurs de confiance.

d'obliger les influenceurs à déclarer leur activité auprès des plateformes qui les hébergent, d'autre part, de rendre visible cette reconnaissance de leur activité d'influence commerciale auprès de l'ensemble des utilisateurs de ces plateformes. Cela ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, ce mécanisme de déclaration et de certification par badge s'apparente tout simplement à la politique de certification en vigueur sur les plateformes en ligne telles que Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter, qui concentrent l'essentiel de l'activité de l'influence commerciale. Ces plateformes attribuent des badges confirmant que le profil appartient bien à une personnalité publique, à un créateur ou à une marque plutôt qu'à un fan ou à un imposteur. Comme vous et moi,

plusieurs vertus. Il permettrait aux internautes de reconnaître distinctement les utilisateurs qui sont amenés à faire de l'influence commerciale,

L'identification des influenceurs commerciaux relève de la responsabilité de chaque réseau social ou plateforme en ligne. C'est un prérequis à leur travail de régulation des contenus illicites. Ce travail sera facilité par l'application du DSA, car les plateformes seront obligées de proposer des fonctionnalités permettant de déclarer le caractère commercial d'une publication et de signaler les contenus illicites. Pour les influenceurs qui s'adressent notamment à un public établi en France, cette proposition de loi facilitera encore davantage leur identification, en rendant obligatoire l'affichage de la mention unique « Publicité ». Toutes ces dispositions sont suffisantes à ce stade pour identifier les comptes des influenceurs.

il n'est prévu aucune sanction dans le cas où lesdites plateformes ne s'exécuteraient pas correctement, alors que cette proposition de loi prévoit de lourdes sanctions contre les influenceurs qui enfreindraient les interdictions mentionnées plus haut. Il importe de responsabiliser les plateformes qui diffusent ces contenus. C'est pourquoi cet amendement prévoit d'appliquer aux plateformes qui acceptent toutes les formes de e-commerce, parfois illicite, illicite, les sanctions prévues pour les fournisseurs de services d'hébergement dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Cela me semble logique. Quel est l'avis de la commission ? L'article 6-1-5 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique ne traite pas des sanctions applicables aux fournisseurs de services d'hébergement, mais de la possibilité pour ces fournisseurs de demander l'annulation des injonctions de retrait qui leur sont transmises. La référence à cet article me semble donc aller à l'inverse de votre objectif, mon cher collègue, qui est d'inciter ces fournisseurs à traiter plus rapidement et plus sérieusement les injonctions de retrait de contenus. Nous aurons d'ailleurs ce débat

Le protocole d'engagements entre l'État et les opérateurs de plateforme en ligne prévoit également la mise à disposition de formations à destination des influenceurs et des agents d'influenceurs. Le secteur est en train de se structurer et, maintenant que le cadre légal est clarifié, chaque acteur doit prendre ses responsabilités. ses responsabilités. Imposer une formation déontologique obligatoire sans conditionner l'exercice de l'activité d'influence commerciale à son octroi s'avérerait inopérant face aux actions déjà menées par le secteur et les pouvoirs publics. La commission est donc défavorable

Au-delà de l'aspect commercial, certaines déclarations d'influenceurs comportent parfois des propos abusifs et dégradants, qui peuvent conduire certaines personnes fragiles à prendre des risques exagérés. On peut penser à la controverse récente sur des promotions relatives au rajeunissement intime ou à certains produits destinés à modifier le teint de la peau. Si ces communications peuvent entrer dans le champ des pratiques commerciales abusives ou trompeuses, il est important que le secteur se dote lui-même d'un arsenal déontologique. Ces règles de déontologie pourraient être définies dans une charte approuvée par l'ensemble des acteurs du secteur. Quel est l'avis cher collègue : nous devons collectivement être plus exigeants à l'égard des plateformes en ligne. Mais leur rôle n'est pas de contrôler le caractère malveillant ou déplacé de leurs publications, mais plutôt de retirer les contenus considérés comme illicites. que vous proposez serait à la fois disproportionnée et contraire au DSA. L'article 4 de ce texte prévoit la signature d'un protocole d'engagements entre l'État et les opérateurs de plateforme en ligne pour améliorer l'efficacité des mécanismes de signalement

collègue : il faut être concis et efficace. Justement, l'intitulé actuel de la proposition de loi

des aliments trop salés ou trop sucrés. Il s'agit d'un vrai problème de santé publique, qui touche les plus défavorisés,

Mais nous ne pourrons pas nous arrêter au milieu du gué. Derrière ce texte se pose toute la question de la publicité, de cette publicité qui induit des modes de consommation et qui, ainsi, oriente la société. Il faudra prendre cette question à bras-le-corps dans les années à venir si nous voulons réorienter

que l'on rend coresponsable des publications. C'est bienvenu, car il n'y avait rien de plus terrible que de voir des agents d'influenceurs faire de l'argent, puis se laver les mains dès qu'il y avait un problème. En revanche, je pense que nous devrons très